a pour objet de tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 28 novembre 2014

et de participer à son élection. Elle a en effet considéré que les militaires, dans les cas où ils pourront être élus, devront pouvoir exercer la plénitude des fonctions liées à ce statut. Compte tenu des élargissements accomplis en termes de repoussement des frontières d'inéligibilité et d'incompatibilité, de deux choses l'une : ou bien les dispositions adoptées permettent aux militaires d'exercer pleinement un mandat politique- dans ce cas, pourquoi ne pas lever toutes les restrictions légales ? -, ou bien la commission est allée trop loin sur l'éligibilité des militaires. Aux États-Unis, la législation en la matière est rigoureuse les membres des forces armées n'ont pas le droit de se présenter à une élection politique ni d'être candidat à aucune autre fonction élective. Le seul assouplissement à cette interdiction est la possibilité pour le secrétaire d'État à la défense d'autoriser les militaires à se présenter à une élection à titre exceptionnel. Toutefois, le secrétaire d'État ne peut pas autoriser le cumul de fonctions : si un militaire est autorisé à participer à une élection, il peut demander à être mis à la retraite s'il remplit les conditions légales

En revanche, on pouvait être militaire en situation de non-activité et éligible. Le Conseil constitutionnel a considéré que cette interdiction avait un caractère général et, partant, disproportionné.

est apparu compatible avec ce principe de neutralité et l'obligation de loyalisme dans les communes de petite taille, où- là aussi, vous le savez mieux que personne -les préoccupations locales l'emportent sur les débats politiques nationaux.

La réflexion de la commission- car nous avons eu de longs débats sur le sujet -est effectivement la suivante : de deux choses l'une, ou bien on autorise les militaires à se présenter, auquel cas on essaie de ne pas leur couper les jambes et les bras et d'en faire des élus à peu près

et il faut savoir qu'au Sénat, au sein de la commission, nous n'étions pas arc-boutés sur l'idée que les militaires puissent participer à la désignation des grands électeurs ou être, eux-mêmes,

d'élus municipaux ! J'ai été maire et je suis encore conseiller municipal d'une commune de 1 500 habitants ; j'ai le sentiment d'avoir autant de légitimité que des collègues d'une commune comme Paris.

Cela m'étonne un peu de la part d'un gouvernement qui entend dépasser les clivages droite-gauche et rassembler tout le monde ! Mais passons sur cet élément anecdotique ... Il me semble qu'un militaire dans un conseil municipal comprenant 15 membres aura beaucoup plus de poids et d'influence qu'un militaire dans un conseil municipal de 50 ou 60 personnes. Ce n'est

le succès sera considérable ou si cette évolution permettra, ici ou là, à un certain nombre de citoyens militaires en activité de s'impliquer dans la vie locale. Nous verrons bien. Mais si cette étape peut amener un questionnement,

tout empêcherait un militaire français de se présenter dans une commune de 9 200 habitants, mais rien n'empêcherait un général allemand disposant d'une maison de campagne en France de se porter candidat dans une commune de 17 000 habitants, d'y être élu et, sans doute, d'en devenir le maire adjoint.

que les grandes catégories que j'ai pu décrire. Néanmoins, cela a été parfaitement rappelé par le rapporteur pour avis de la commission des lois, ainsi que par le président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, le Conseil constitutionnel, lui-même, nous invite à nous orienter vers les seuils.

pour une autre position administrative et évoluer d'une position d'activité à une position de détachement, ce qui est parfaitement possible. Il n'y a donc aucun ostracisme d'aucune sorte vis-à-vis des militaires et je suis la première convaincue que

même lorsque ceux-ci sont titulaires d'un mandat local. Il tend à rétablir l'interdiction, introduite à l'Assemblée nationale,

les priver de la possibilité de se présenter à l'élection des délégués des conseils municipaux en vue de l'élection sénatoriale, et de voter à cette élection.

Ces principes font effectivement obstacle à ce que les militaires en activité sollicitent le suffrage des autres conseillers municipaux, en s'inscrivant sur des listes de grands électeurs. Cette démarche suppose un engagement partisan avéré, d'autant plus marqué qu'il s'agit d'un collège électoral restreint.

Tout d'abord, il vise à étendre, aux fonctions de maire délégué et d'adjoint au maire délégué, l'incompatibilité prévue avec les fonctions de maire et d'adjoint au maire. Sauf accord de l'ensemble des communes regroupées, la création de communes déléguées reprenant les noms et limites territoriales des anciennes communes intervient automatiquement en cas de création d'une commune nouvelle. Le nombre de ces communes a donc crû au cours des dernières années, et devrait continuer d'augmenter. La plupart des communes concernées sont d'une taille réduite. les maires délégués disposent de pouvoirs étendus : ils sont officiers d'état civil, officiers de police judiciaire ; ils peuvent être chargés de l'exécution des lois et règlements de police, recevoir des délégations du maire ; ils exercent également des fonctions d'adjoint au maire de la commune nouvelle. Ces différentes missions peuvent être lourdes. Dans cette mesure, elles sont, tout comme les missions de maire ou d'adjoint au maire, incompatibles avec l'exigence constitutionnelle de disponibilité qui pèse, à nouveau, sur les militaires en activité. En outre, cet amendement tend à harmoniser les dispositions relatives à la participation des militaires en position d'activité aux structures intercommunales, précisant que les incompatibilités applicables pour l'élection des délégués des syndicats de communes sont, notamment, celles qui sont prévues pour les élections au conseil communautaire par l'article L. 46 du code électoral. À défaut, en effet, s'appliqueraient pour les syndicats de communes les seules règles d'incompatibilité applicables aux communes, soit un seuil démographique de 9 000 habitants apprécié à l'échelle de la commune, et non,

Rien ne justifierait une telle différence de régime ! Il serait donc incohérent de permettre à un militaire en position d'activité de siéger dans l'organe délibérant d'un EPCI d'une certaine taille, dès lors qu'il réside dans une commune membre de moins de 9 000 habitants

Je me demande donc dans quelle mesure- et je me tourne, pour cela, vers les éminents membres de la commission des lois -il n'y aurait pas nécessité de recourir à un support constitutionnel pour garantir ce droit. De surcroît, du fait d'empêcher un militaire d'être désigné délégué, au titre des citoyens désignés par le conseil municipal dans les communes de plus de 30 000 habitants, le Conseil constitutionnel contrôle toute dérogation entre la qualité

aux militaires de participer à la désignation des députés, pour la raison très simple que le suffrage universel est direct. Les militaires ne souffrent évidemment d'aucune forme d'ostracisme par rapport aux autres citoyens.

Sans vouloir prolonger inutilement ce débat, permettez-moi de vous dire que certains propos m'ont choquée. On ne peut pas parler de déni de démocratie, comme je l'ai entendu tout à l'heure. Si ! Il s'agit de la stricte application de nos règles constitutionnelles.

! -, un monde à la fois d'expérience, de sensibilité et de très grand respect des grandes valeurs qui fondent la République et, en ce qui me concerne, qui fondent le gaullisme. L'amendement n° 78 vise à sécuriser l'exercice du mandat municipal des militaires. Le code général des collectivités territoriales prévoit que tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir l'une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. En raison de sa disponibilité dans l'armée, un militaire peut être amené à ne pas pouvoir exercer certaines fonctions, notamment celles d'assesseur lors d'une élection

Yung, sur l'article. Nous abordons maintenant un chapitre important, concernant la cyberdéfense. Je veux souligner précisément l'importance de traiter ces questions, y compris dans le cadre de la loi de programmation militaire. L'enjeu est de taille. Partout, dans le monde, les États se dotent des outils

C'est pourquoi la France doit se doter des ressources technologiques et humaines nécessaires. C'est ce que prévoit le présent projet de loi, par une augmentation des effectifs de cyberdéfense à hauteur de 1 000 personnes ainsi qu'à travers un budget de 1,6 milliard d'euros, hors masse salariale. Mais notre réponse doit aussi être juridique. Tel est aussi l'objet de l'article

et les débordements, le principe de précaution s'appliquera, puisque les activités de l'ANSSI seront contrôlées par l'Autorité de régulation des communications électroniques

Mme la ministre. Cet amendement a pour objet de simplifier les dispositions applicables au recours juridictionnel à disposition de l'ARCEP en cas de méconnaissance d'une injonction adressée à l'ANSSI. Votre commission a souhaité garantir l'effectivité du contrôle de l'ARCEP sur la mise en oeuvre des nouveaux outils de détection dont la loi va doter l'ANSSI, en lui ouvrant une voie de recours spécial devant la formation spécialisée du Conseil d'État. Pourtant, une telle voie de recours me semble inappropriée. Tout d'abord, je veux souligner que l'ANSSI ne manquera pas de déférer aux injonctions de l'ARCEP et rappeler que le droit au recours existe, même sans texte. L'ARCEP en dispose, même si la loi ne le prévoyait pas La loi peut, certes, rappeler que l'ARCEP peut saisir le Conseil d'État. Le présent amendement ne remet pas cette dimension en cause. ce qui paraît tout à fait inapproprié, c'est de confier ce contentieux à la formation spécialisée du Conseil d'État, dont ce n'est pas le rôle. La loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement a créé, en effet, au sein du Conseil d'État, cette formation spécialisée, dans un but bien précis, qui est de connaître des litiges relatifs à l'utilisation des techniques de recueil de renseignements et à l'exercice du droit d'accès indirect aux fichiers de renseignement. La justification d'une telle création repose évidemment sur la spécificité des activités de renseignement couvertes par le secret, ainsi que par le caractère intrusif des techniques mises en oeuvre, compte tenu des risques d'atteinte à la vie privée. Or les dispositifs techniques mentionnés à l'article 19 répondent à une logique tout à fait autre, puisqu'ils n'impliquent pas, par eux-mêmes, d'atteinte à la vie privée ni au secret des correspondances. C'est ce qui explique que le contrôle de leur mise en oeuvre soit confié à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, et non pas à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

au-delà de sa raison d'être, c'est-à-dire les activités de renseignement, ferait perdre sa cohérence à cette voie de droit tout à fait spécifique et fragiliserait le régime procédural qui lui est attaché. Par ailleurs, j'ajoute que, devant les juridictions supranationales, le caractère très particulier de son champ d'intervention est un argument important. Les juridictions de droit commun pourront, quoi qu'il en soit, être saisies et, à ce titre, le présent amendement maintient bien la possibilité pour l'ARCEP de saisir le Conseil d'État, mais en formation ordinaire, et de faire usage, si nécessaire, des procédures d'urgence ouvertes devant le juge administratif.

Ainsi, le seul fait que le contentieux propre à la mise en oeuvre des dispositifs techniques puisse concerner des informations classifiées ne peut à lui seul justifier un recours devant la formation spécialisée du Conseil d'État, sauf à vouloir fragiliser le rôle de la Commission consultative du secret de la défense nationale. C'est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir accepter la modification

d'abord, en lui donnant accès au dispositif de traçabilité des données et en lui permettant d'être assistée par des experts habilités.

Restreindre les catégories de données techniques susceptibles d'être ainsi recueillies aurait pour effet de limiter les capacités de l'ANSSI à analyser le mode opératoire d'un attaquant, sans pour autant renforcer le droit au respect de la vie privée qui n'est pas, en soi, affecté par cette analyse. l'expérience montre que les techniques d'attaque évoluent sans cesse, en tout cas extrêmement rapidement. Le risque existe donc que des données qui auraient été préalablement préalablement définies par grandes catégories dans un décret ne soient plus celles qu'il serait pertinent de recueillir. Dans ces conditions, le recours à un décret en Conseil d'État pour définir la nature la nature des données conservées par l'ANSSI dans le cadre spécifique de la mise en détection d'un équipement qui aurait été infecté par un attaquant me paraît tout à fait contre-productif. En revanche, un décret en Conseil d'État pourrait, conformément au souhait exprimé par la commission, préciser les modalités d'application de ce dispositif

la définition précise des catégories de données, madame la ministre, est une des conditions permettant au Conseil constitutionnel de considérer que la collecte et la conservation par les opérateurs ne portent pas une atteinte disproportionnée au secret des correspondances et au respect de la vie privée. donc les mêmes arguments qui nous ont conduits à préciser que le décret devait inclure les catégories de données que l'ANSSI pouvait essayer de saisir. Cette simple précision

il convient de définir les catégories de données que l'ANSSI est autorisée à collecter lorsqu'elle met en oeuvre des sondes de détection sur les réseaux ou sur les serveurs des opérateurs,

en confiant un rôle tant aux opérateurs de communication électronique et de téléphonie qu'à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Je veux souligner le travail

nos deux commissions- je pense, par exemple, à la clarification des obligations des opérateurs de communication. Nous avons conforté le contrôle de l'ARCEP en créant un lien de contrôle juridique avec l'ANSSI. Nous avons étendu aux opérateurs de services essentiels le périmètre de la détection et de la protection. Je veux remercier le Gouvernement d'avoir accepté la plupart de nos amendements. Il nous reste un petit point de désaccord, mais je pense que nous aurons l'occasion de trouver, avec nos collègues de l'Assemblée nationale, une rédaction

nous proposions que ce décret en Conseil d'État examine les modalités d'un renforcement de garanties, dont nous ne doutons pas

de procéder à des contrôles sur les campagnes d'essais. Le dispositif retenu par l'Assemblée nationale est fondé sur un régime de déclaration préalable des campagnes d'essais de matériel de renseignement auprès de la

Ce contrôle se traduit par la possibilité, pour la CNCTR, d'obtenir, sur sa demande, communication du registre qui recense les opérations techniques effectuées.

aurait pour effet d'entretenir une confusion entre la mise en oeuvre des techniques de renseignement, qui peut être soumise à des contrôles approfondis par la CNCTR, et les simples essais de matériel de renseignement qui doivent répondre à un contrôle moins poussé. Il y aurait donc un paradoxe à prévoir un contrôle sur place pour de simples essais de matériel, alors même que le législateur a a exclu tout récemment cette possibilité dans le cadre de la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme en ce qui concerne la mise en oeuvre par les armées de mesures de surveillance peu attentatoires à la vie privée, c'est-à-dire relevant de techniques dites de « hertzien ouvert ». En effet, les unités des armées autorisées à mettre en oeuvre de telles mesures ne sont pas soumises à un contrôle sur place de la CNCTR, dernière étant uniquement informée du champ et de la nature des mesures de surveillance hertzienne, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 21 octobre 2016 et à l'avis de l'assemblée générale du Conseil d'État du 15 juin 2017.

Pour l'ensemble de ses raisons, je vous demanderai de bien vouloir revenir sur la disposition votée en commission. Quel est l'avis de la commission ? La commission

la stricte limite nécessaire, raison pour laquelle ce contrôle sur place nous semblait important. La commission a décidé de s'en remettre à la sagesse du Sénat.

Cet amendement répond à une double nécessité. Tout d'abord, il convient de permettre aux services de n'engager qu'avec discernement la surveillance des communications d'un individu.

La séparation étanche entre surveillance des communications nationales et internationales pose des difficultés que l'évolution de la menace met au jour.

pour permettre un droit de suite quand une personne menaçante quitte notre sol. Mais il n'est pas possible d'exploiter les données légalement recueillies au titre de la surveillance des communications internationales pour apprécier la menace que présente un résident français en France du fait de ses liens hors du territoire national. est donc difficilement compréhensible que l'on se coupe ainsi de données légalement recueillies. Par exemple, un résident français qui planifierait un attentat depuis le Yémen peut être surveillé.

messieurs les sénateurs, de permettre simplement une utilisation plus rationnelle des données légalement recueillies dans le cadre de la surveillance des communications internationale. Nous ne donnons pas aux services de nouveaux moyens de collecte ni ne modifions en profondeur les équilibres retenus en 2015. La levée de doute prendra la forme d'une vérification ponctuelle sur les données de connexion légalement interceptées dans le cadre de la surveillance des communications internationales. Il s'agit d'opérations très rapides, non répétées et susceptibles de mettre en évidence un graphe relationnel ou la présence à l'étranger d'une personne, qui pourra alors être surveillée si elle présente une menace. Dès que la vérification fera apparaître la nécessité d'une surveillance, l'exploitation des communications ne pourra être poursuivie que les techniques de renseignement inscrites dans la loi de 2015, dans le respect des garanties procédurales qui les entourent. Nous voulons toutefois aller plus loin dans deux cas très particuliers. D'abord, pour prévenir des menaces terroristes urgentes, les services doivent pouvoir recourir à un tamis plus fin, permettant une orientation plus rapide de leurs investigations. Il est donc prévu que, dans ce cas, les vérifications ponctuelles puissent porter sur des correspondances, avec une obligation de traçabilité renforcée, dans la mesure où des

celles qui sont susceptibles de mettre en cause l'indépendance nationale ou les intérêts de la défense nationale, il faut aussi que les vérifications ponctuelles puissent porter sur les correspondances. La démarche proposée est très différente : il ne s'agit pas de mettre en évidence la menace ou la vulnérabilité que présente un individu, mais des marqueurs techniques de flux malveillants circulant entre des machines victimes ou relais de l'attaque.

Cet amendement comporte un second volet : pour mieux prendre en compte les menaces transnationales, nous prévoyons deux mesures. Nous voulons d'abord permettre l'exploitation des données d'un identifiant technique rattachable au territoire national interceptées dans le cadre de la surveillance des communications internationales, alors même que son utilisateur est en France. Aujourd'hui, ce n'est pas possible et c'est une faille importante. Cette surveillance ne pourra être demandée que pour la promotion et la défense de certains des intérêts fondamentaux de la Nation, ceux que compromettent des menaces transnationales. Elle relèvera d'une autorisation individuelle du Premier ministre, après avis de la CNCTR. La même démarche d'adaptation de la frontière entre les régimes applicables en France et à l'étranger conduit à prévoir une mesure de moindre portée. Il s'agit de mettre fin à une situation peu cohérente résultant de la rédaction de la loi, afin que certaines techniques de renseignement autorisées sur le territoire national puissent puissent permettre l'exploitation des données strictement correspondantes interceptées dans le cadre de la surveillance des communications internationales. Ainsi, les interceptions de sécurité donneraient accès pour trente jours au flux des communications mixtes, vers ou depuis l'étranger, les demandes de « fadettes » permettraient d'obtenir un double relevé de données de connexions nationales et internationales, sur une durée bornée à un an.

qui utilise les moyens de communication et de télécommunication, soit avec des numéros français commençant par 33, soit avec des numéros étrangers, mais opérant depuis la France, il faut évidemment donner à nos services tous les moyens pour renforcer la surveillance électronique de ces communications. Ensuite, nous nous sommes

est motivé par le constat que la menace est transnationale, comme Mme la ministre l'a fort bien expliqué, et qu'il existe une nécessité opérationnelle d'exploiter des données légalement recueillies au titre de la surveillance des communications internationales

que les membres de la délégation pourront se déplacer directement sur le site où ces agents opèrent, de manière à ne pas mettre en péril leur anonymat, autrement dit leur couverture. Mais c'est justement le contraire qui risque de se produire ! Cet article prévoit en effet l'audition d'agents sur le lieu même de leur action. Une telle mesure est hautement susceptible d'exposer leur identité. La venue d'un groupe de députés ou de sénateurs,

l'objet initial de cette délégation parlementaire est « le suivi de l'activité générale des moyens des services de renseignement ». En aucun cas il n'est fait mention d'une forme de contrôle généralisé.

ainsi libellé : La parole est à Mme la ministre. Cet amendement a pour objet d'écarter la possibilité d'un contrôle de la délégation parlementaire au renseignement sur l'ensemble de l'activité des services de renseignement. La loi du 9 octobre 2007, qui a créé la délégation parlementaire au renseignement, permet l'information du Parlement sur l'activité des services de renseignement selon les exigences propres à toute démocratie. Ses possibilités d'audition et d'obtention de documents ont été accrues bien légitimement, à l'occasion d'évolutions législatives successives, la dernière ayant eu lieu en 2015. Le Gouvernement a naturellement à coeur d'établir et d'entretenir une relation de travail dense entre les services de renseignement et la délégation parlementaire au renseignement. Toutefois, l'article dont nous discutons introduit à notre sens un véritable bouleversement, qui pose d'importantes difficultés juridiques et opérationnelles. Pour l'exercice de ses missions, la délégation reçoit des informations sur le budget, l'activité générale et l'organisation des services, mais pas sur l'activité opérationnelle des services. Or le présent article remet profondément en cause cet équilibre, en reconnaissant un droit à l'information sur l'ensemble des pans pans de l'activité des services de renseignement, qu'il s'agisse d'informations relatives aux procédures et aux méthodes opérationnelles, des échanges avec les services étrangers partenaires ou encore d'informations, comme cela a été rappelé à l'instant, concernant les agents des services spécialisés, qui sont pourtant protégés par le droit au respect de l'anonymat. Il existe donc à ce titre un véritable risque d'atteinte au principe de séparation des pouvoirs et aux prérogatives constitutionnellement garanties au pouvoir exécutif. Le présent article ouvre en effet la possibilité d'une information de la DPR sur les opérations en cours, alors même que le Conseil constitutionnel juge que le contrôle opéré par le Parlement ne peut concerner de telles opérations. ailleurs, cet article vise à conférer à la délégation parlementaire au renseignement une faculté de supervision de l'action des services de renseignement qui ne respecte pas la délimitation du rôle du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, qui a été consacrée par la jurisprudence constitutionnelle, lorsque le pouvoir exécutif intervient dans le cadre de sa mission de défense des intérêts fondamentaux de la Nation. En outre, un tel droit à l'information sur l'ensemble des pans de l'activité des services de renseignement est de nature à entraver l'efficacité opérationnelle des services et à mettre en péril leur sécurité opérationnelle, ainsi que celle de leurs agents. L'article tend à fragiliser les méthodes de travail et les modalités d'action des services de renseignement, qui sont fondées sur le principe de cloisonnement de l'information. Ce cloisonnement se traduit par l'octroi d'habilitations et ce que l'on appelle le « besoin d'en connaître », qui restreignent l'accès à l'information au sein même des services. La sécurité des personnels et des opérations est ainsi assurée, aucun agent n'ayant accès à l'ensemble des informations détenues par le service.

alors que l'accord exprès d'un partenaire est requis pour mettre à disposition d'un tiers des informations qu'il a partagées. Par ailleurs, cet article confère à la DPR, sans aucunement l'encadrer, un droit nouveau : celui de se rendre sur le site d'un service de renseignement et d'y auditionner tout le personnel.

qui ont précisément visé à protéger de façon systématique l'anonymat des agents des services de renseignement. Par ailleurs, elle contrevient aux dispositions de l'article 20 de la Constitution aux termes duquel le Gouvernement dispose de l'administration. Je ne l'ignore pas, les promoteurs de cet amendement invoquent des exemples étrangers. Oui ! Mais on ne peut isoler des dispositions de contrôle des services étrangers des prérogatives de ces derniers ni du contexte politique et juridique de chaque pays. Chaque système repose sur un équilibre différent. On ne peut importer, comme cela, certains éléments parcellaires provenant d'autres législations, sans repenser l'ensemble.

Je l'ai indiqué tout à l'heure, ce texte devrait faire l'objet, en 2020, après cinq années de mise en oeuvre, d'une évaluation par le Parlement. C'est donc dans ce cadre, ou à l'occasion de l'examen d'un vecteur législatif dédié, qu'il me semble plus propice d'examiner, conformément à une démarche de concertation entre les services concernés et le Parlement, la question de la réévaluation des pouvoirs de la délégation parlementaire au renseignement, à l'aune de l'expérience de la mise en oeuvre des dispositions récentes qui les ont renforcés. Je ne doute pas qu'une telle évolution sera de nature à consolider la relation nécessaire de confiance avec les services de renseignement, que le législateur a souhaité instaurer lors de la création de la délégation parlementaire au renseignement en 2007. Inversement, il serait difficilement compréhensible que, sur un sujet aussi important et aussi sensible, qui touche au coeur de la souveraineté de notre pays, un amendement non concerté avec le Gouvernement vienne porter atteinte au bon fonctionnement de nos services de renseignement et à la sécurité de leurs opérations et de leurs agents. Je vous invite donc, mesdames, messieurs les sénateurs, à adopter le présent amendement,

Celui-ci a été adopté par nos deux commissions. Il résulte des recommandations délibérées au sein de la délégation parlementaire au renseignement, lorsqu'elle a adopté son rapport au mois d'avril dernier. rapport au mois d'avril dernier. Il ne s'agit nullement de nous substituer au pouvoir exécutif. Tout votre raisonnement sur la séparation des pouvoirs est parfaitement hors de propos, puisque vous parlez de séparation des pouvoirs, vous ne contesterez pas que l'article XV de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, selon « la Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration », doit s'appliquer à toutes les fonctions de l'État, y compris à la fonction de renseignement. évidemment s'y appliquer dans des conditions particulières, car il ne s'agit en aucun cas de fragiliser ni des opérations en cours, ni la coopération avec des services étrangers, ni des agents ou des sources

au renforcement des pouvoirs de contrôle du Parlement. Nous voulons nous aussi contribuer à ce renforcement, mais nous voulons le faire avec discernement. C'est la raison pour laquelle, en nous inspirant en effet des exemples étrangers, sans pour autant copier la constitution américaine, nous voulons mettre à niveau le contrôle parlementaire et permettre à notre délégation parlementaire au renseignement de franchir ainsi un palier dans l'exercice de sa responsabilité au nom de la représentation nationale, en prévoyant que, au lieu d'être destinataire d'une liste limitative de documents prévus par la loi,

pourraient compromettre la sécurité et l'efficacité de nos services. C'est un très bon

pour les intérêts fondamentaux de la Nation soit pleinement respectée, le Gouvernement conservant la clé de l'information qu'il communique. Quant à la possibilité, reconnue

Selon moi, votre réponse participe d'une méfiance à l'égard de la représentation nationale. Pour notre part, nous exprimons notre confiance à l'égard des services de renseignement. Mais la confiance n'exclut pas le contrôle ! Ils vont de pair : le contrôle s'effectuera dans un esprit de responsabilité, et les dispositions que nous avons prévues permettront à nos services de renseignement d'avoir la garantie qu'il n'y aura pour eux aucun risque. je vous le rappelle, la délégation parlementaire au renseignement, du fait de la loi elle-même, a accès aux secrets de la défense nationale, et ses membres sont assujettis à ce secret. On ne peut retenir l'idée étonnante

la saisine : « Cet article encourt, sinon la censure, du moins de strictes réserves d'interprétation en ce qu'il enfreint le principe de la séparation des pouvoirs et, en particulier, l'exclusivité des responsabilités du Président de la République et du Premier ministre en matière de défense nationale. Tout d'abord, la désignation au sein de la commission n'est pas subordonnée à une habilitation de niveau Très Secret-Défense. [ ...] Ensuite, la commission reçoit communication de l'état des dépenses se rattachant à des opérations en cours, ce qui est susceptible de compromettre la sécurité de celles-ci.

de la décision du Conseil constitutionnel : « Considérant que, selon les sénateurs requérants, cette disposition méconnaîtrait les prérogatives du Président de la République et du Premier ministre dans la conduite des affaires relevant de la défense nationale et mettrait en péril la sécurité des opérations des services secrets " ; considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 5 de la Constitution, le Président de la République " est garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités qu'en vertu de son article 15, il est " le chef des Armées " ; que son article 21 dispose que le Premier ministre " est responsable de la Défense nationale " ; qu'aux termes de son article 35, le Parlement autorise la déclaration de guerre ; qu'en application de ses articles 34 et 47, le Parlement vote, à l'occasion de l'adoption des lois de finances, les crédits nécessaires à la défense nationale ; considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions constitutionnelles précitées que, s'il appartient au Parlement d'autoriser la déclaration de guerre, de voter les crédits nécessaires à la défense nationale et de contrôler l'usage qui en a été fait, il ne saurait en revanche, en la matière, intervenir dans la réalisation d'opérations en cours ; qu'il y a lieu, dès lors, de déclarer contraires à la Constitution les dispositions » de l'article instaurant la commission de vérification des fonds spéciaux. de la méthode, monsieur le président, je ne suis pas constitutionnaliste ; en outre, je vous l'accorde, nous étions en 2001, c'est-à-dire à la fin du XXsiècle, et nous sommes aujourd'hui en 2018. Entre-temps, la législation sur le renseignement s'est évidemment considérablement enrichie. Mais la Constitution, elle, reste fondamentalement la même, même si, là aussi, quelques évolutions ont pu intervenir. S'agissant de la méthode, donc, très sincèrement que ces matières sont suffisamment sensibles pour que nous prenions le temps de les examiner sereinement, sur le fond.

de ces échanges d'arguments, vifs et passionnés- il s'agit quand même de matières sérieuses ! -, envisager de reprendre ces questions dans un autre cadre, en prenant le temps, car- je le redis -il ne s'agit nullement de contrarier le contrôle parlementaire ? Et je ne souscris pas à certains propos qui ont été tenus tout à l'heure, selon lesquels ce gouvernement serait défavorable au contrôle exercé par le Parlement. C'est le contraire

par le président Bas. Tout d'abord, vous évoquez cette décision du Conseil constitutionnel de 2001 ; elle date tout de même d'un certain nombre d'années. Depuis, la notion de contrôle parlementaire a beaucoup évolué, y compris dans la jurisprudence du Conseil du Conseil constitutionnel. Ensuite, je vous redis que nous vous tendons la main- je l'ai dit dans mon propos liminaire. Il n'y a donc aucune volonté d'affrontement, simplement la volonté de doter le Parlement des moyens nécessaires à l'évaluation des opérations de renseignement,

sont en droit de recevoir un retour sur les engagements d'effectifs et de crédits mis en oeuvre. J'ai l'honneur de siéger, auprès du président Bas, au sein de la DPR. Je peux vous dire,

la commission de vérification des fonds spéciaux, qui est une émanation de la DPR, se rend dans un certain nombre de pays et fait son travail de la manière la plus discrète possible.

à tous ces hommes et à toutes ces femmes qui, dans l'ombre, dans des pays parfois très agités, remplissent leur mission au péril de leur vie.

depuis 2001. Il y a vraiment lieu de contrôler le plus efficacement possible, mais sans que la confiance soit rompue avec

Premièrement, l'opacité autour de la nature du fichier BIOPEX est totale. Si la sécurité nationale peut justifier un accès limité, il faut quand même prendre la mesure de ce fichier

Ceci nous interroge d'autant plus que les activités de nos militaires ne se bornent pas à la lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, les risques de « dérapages » sont pourtant limités, puisque le fichier BIOPEX ne concerne que les combattants décédés, lors d'actions de combat, ou capturés par les forces armées. Il s'agit donc,, d'identifier une personne et de faire la preuve de sa culpabilité. Mais la réforme proposée modifie diamétralement le dispositif. Il ne s'agira plus d'identifier et de confondre, mais de tout faire reposer sur l'intuition de nos militaires. La protection des militaires est une priorité absolue, mais j'ai du mal à voir en quoi cet article permet Soit le dispositif est pleinement utilisé, et l'on va vers un fichage généralisé susceptible de créer des troubles ; soit le fichage se concentre sur des suspects déjà établis dont les services de renseignement s'occupent déjà. La seule garantie apportée par le texte, à savoir la mention des motifs « précis et sérieux », est bien floue pour être efficace. Faudrait-il considérer ceux que certains appellent des agitateurs publics comme constituant une menace « précise et sérieuse »

un risque que l'armée française passe pour une force d'occupation plus que de protection. Et nous supposons que la sécurité des militaires serait ébranlée tout autant par un rejet de la population que par l'impossibilité de prélever à tout-va des données pour BIOPEX. ces raisons, nous vous proposons la suppression de cet article.

Selon le Conseil d'État, cet article s'inscrit dans le cadre des conventions de Genève. Ces dernières sont elles-mêmes fondées sur la distinction entre civil et soldat. Le droit international humanitaire ne reconnaît donc pas d'autre catégorie Or, dans les conflits actuels, les combattants ne portent pas forcément d'uniforme. Ils peuvent être en civil le jour, et combattants la nuit. Je me pose donc la question suivante : à quel statut correspond la catégorie des « personnes dont il existe des raisons précises et sérieuses de penser qu'elles présentent une menace » ? La rédaction de l'article ne résout pas cette difficulté. Les personnes visées ne sont considérées ni comme combattantes, ni comme prisonnières, ni comme civiles. Ma question rejoint celle qui vient d'être posée ; elle est simple : en cas de refus de l'individu, sur quel droit peut s'appuyer notre soldat pour le soumettre au prélèvement ? considérer les conséquences de l'application de cette mesure sur les relations avec la population locale. En opérations extérieures, notre armée essaie, dans la mesure du possible, de se mêler à la population, ce qui n'est pas le cas d'autres armées comme l'armée américaine ou l'armée chinoise. Je crains que de tels prélèvements conduisent à une suspicion généralisée de la part de la population ; une telle suspicion ne peut produire qu'une défiance à l'encontre des forces françaises. Cet ajout au code de la défense ouvre donc plus de questions qu'il n'apporte de réponses. C'est pourquoi je propose sa suppression.

attendue par nos militaires, c'est certainement celle-là : la possibilité d'opérer un certain nombre de prélèvements à la suite d'arrestations de

un IED, autrement dit sur une mine artisanale. Admis à l'hôpital Percy, il avait définitivement perdu un bras, une jambe et les deux yeux. Croyez-moi : à ce moment-là, on ne regarde pas le code pour savoir si les mesures que l'on prend sont adéquates.

un terrorisme qui prend plusieurs visages. Je souhaite que vous soyez le plus grand nombre à aller voir sur place

Selon le rapport annexé à la présente LPM, certains partenariats stratégiques ont acquis une telle importance qu'ils sont mentionnés au titre de la fonction d'« intervention », au même titre que nos engagements auprès de l'OTAN. Face à la prolifération d'engagements et de coopérations, même informels, qui ont des implications pour la défense nationale, il nous semble important de réaliser un état des lieux bisannuel des partenariats existants, de leur adéquation avec nos intérêts nationaux et de leur compatibilité avec les moyens alloués à nos forces dans le cadre de la LPM. Il nous semble également essentiel que l'information du Parlement soit renforcée et que la représentation nationale puisse débattre des implications de ces partenariats, sans bien sûr s'immiscer dans les prérogatives de l'exécutif en la matière. Quel est l'avis de

Ces commissaires, déjà importants lorsque les entreprises exportatrices étaient publiques, sont aujourd'hui vitaux alors que les prestataires sont privés. sont privés. Nous souhaitons renforcer le contrôle de l'État sur ces entreprises, marquant la spécificité de l'industrie d'armement. Car, comme je l'ai déjà évoqué, cette dernière est politique avant d'être économique. d'abord, car l'exportation d'armements est, qu'on la condamne ou qu'on l'approuve, un outil de diplomatie important, comme l'a montré l'épisode de la vente des Mistral à la Russie, puis finalement à l'Égypte, avec financement saoudien. ensuite, car, au-delà du profit, c'est toute une stratégie industrielle qui doit être discutée. Comment la France a-t-elle pu sacrifier 44 000 emplois entre 2008 et 2013, tout en montant en charge en matière d'exportations ? Comment expliquer que, avec 10 % à 20 % de chiffre d'affaires, des entreprises exportatrices consacrées à la recherche et au développement présentent une part si faible d'emplois convertis dans le civil ? politique enfin, car la nature même des matériels concernés fait de l'armement une industrie spécifique qui doit relever du contrôle politique. Sans cela, il y a toujours le risque que la recherche absolue de profits n'entre en confrontation directe avec l'ambition de la France de lutter contre la prolifération des armes conventionnelles. Quel

Cela passe par une réforme interne de l'organisation, afin d'enrayer tout blocage. Il est essentiel de mener une politique claire vis-à-vis des États qui se soustraient à l'autorité des Nations unies. Nations unies. L'arrêt de la vente d'armes à ces pays serait à la fois un fort message politique et une sécurité pour la France elle-même. La crainte est que la France perde toute crédibilité à condamner des opérations extérieures illégales alors que ses propres armes sont parfois sur le terrain. Nous pensons, par exemple, au Yémen, où des armes françaises pourraient être impliquées. Madame la ministre, nous avons bien entendu votre intervention du 9 février dernier, expliquant que les armes françaises vendues à l'Arabie Saoudite n'étaient « pas censées être utilisées au Yémen au Yémen ». Notre amendement va donc dans votre sens. Si nous ne vendons plus à des pays intervenant sans mandat de l'ONU et dont les pratiques constituent de graves atteintes aux droits humains, les armes françaises ne se retrouveront plus associées à de véritables crises humanitaires. crises humanitaires. J'ajoute que nous avons été quelque peu indignés lorsque le porte-parole du Gouvernement a déclaré que la vente d'armes françaises à l'Arabie Saoudite était « un intérêt clair pour l'industrie française ».

De fait, l'adoption de notre amendement ne ferait que légitimer l'ONU dans son action pour la paix. Quel est l'avis de la commission ? En

Christine Prunaud. Apparue pour la première fois dans le cadre de la LPM de 1996, l'information au Parlement sur les exportations d'armes s'est généralisée lors de l'examen du projet de loi de programmation militaire de 2013. Cependant, aujourd'hui, les limites du rapport sont régulièrement observées. Tout d'abord, on note une certaine confidentialité du rapport annuel faute de débat au Parlement sur son contenu. Ensuite, il manque un espace de contrôle, puisque ce rapport ne fait même pas l'objet d'un vote, ne serait-ce que symbolique, permettant une prise de position du Parlement sur la politique menée en matière d'exportation d'armements. Enfin, l'opacité est totale, puisqu'il manque à ce rapport de nombreux éléments susceptibles d'éclairer la représentation nationale.

Je dis « enfin », car il faut quand même rappeler que ce projet de loi a été porté par Mme Michèle Alliot-Marie. Plus de dix ans après son adoption par l'Assemblée nationale et cinq ans après son adoption par le Sénat, ce texte n'est toujours pas arrivé au bout de son processus. Pourtant, il nous semble qu'on peut difficilement s'opposer à un texte voté par deux majorités différentes et visant seulement à créer un délit d'infraction aux embargos, ce qui semble relever du bon sens. Cet amendement comporte deux enjeux spécifiques. Le premier, qui concerne l'adoption de telles dispositions, viendra légitimer les organisations internationales, en l'espèce l'Union européenne, l'ONU et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. En effet, il apparaît difficile de se satisfaire du fait que des embargos décidés par la communauté internationale ne soient pas respectés. J'ajouterai par ailleurs que, du fait des insuffisances du rapport français annuel sur les exportations d'armement, rien n'indique aujourd'hui que les livraisons de matériel, par exemple en Côte d'Ivoire, en Chine, en Biélorussie, en Russie ou encore en République démocratique du Congo, ne tombent pas sous le coup des embargos applicables à ces pays. Le second enjeu est, bien évidemment, humanitaire. Il s'agit de ne pas oublier que, derrière ces embargos, se cache bien souvent la volonté de limiter les risques d'une explosion armée sur des territoires instables, pouvant à tout moment déboucher sur de vraies crises humanitaires. Une nouvelle fois, ces dispositions s'inscrivent pleinement dans le droit international, que ce soit le traité sur le commerce des armes ou la résolution

Mon cher collègue, vous avez tout à fait raison s'agissant de la procédure législative. Effectivement, ce texte a fait l'objet de deux votes successifs : l'un au Sénat, en 2007, et un autre à l'Assemblée nationale, en 2016.

si vous en étiez d'accord, de poursuivre le travail et de retirer votre amendement. Nous retrouverons ce texte ultérieurement. Monsieur